La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après l'engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

trop restrictive et présentant une connotation qualitative difficile à apprécier, est remplacée par celle d'« équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées » par le CFA. Cette modification permet de renforcer la capacité de versement de fonds par les entreprises pour développer l'offre de formation de tous les types de CFA, y compris des CFA internes aux entreprises.

Ces centres s'attachent à dispenser une formation fondée sur un triple projet : premièrement, garantir une formation sportive de haut niveau permettant l'accès à une carrière professionnelle ; deuxièmement, assurer une formation humaine fondée sur un cursus d'enseignement permettant d'accéder à des études supérieures,

correspondant au hors-quota, ou barème. Le montant considéré représentait 23 % de la taxe d'apprentissage due. Depuis 2014, seuls les diplômes professionnels délivrés par le ministère des sports permettent aux centres de formation de percevoir une partie de la taxe d'apprentissage.

au même titre que les établissements dispensant des formations initiales technologiques et professionnelles conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

que seuls les établissements d'enseignement supérieur gérés par des organismes sans but lucratif sont éligibles au solde de la taxe d'apprentissage. D'ailleurs, tel est le cas aujourd'hui. Il me semble cohérent d'introduire la même précision au sujet des établissements du

de lever les stéréotypes liés aux formations technologiques et professionnelles, de rapprocher les mondes de l'école et de l'entreprise, grâce à l'organisation de rencontres et d'échanges, et de mettre à disposition des ressources pour que les jeunes s'informent sur leurs possibilités de formation.

s'être entretenue avec la commission de la culture, notre commission a abaissé le taux en question de 20 % à 10 %. Ce faisant, elle est revenue à la proposition initiale du Gouvernement, afin de ne pas diluer de manière excessive les financements dédiés aux établissements éligibles à la taxe d'apprentissage.

un peu moins de 11 millions d'euros au titre du hors-quota, soit 2,6 % des sommes affectées aux organismes et établissements éligibles. Un plafond de 10 % ne me semble pas de nature à mettre en péril les financements dont bénéficient ces associations.

il convient de supprimer également les dispositions en vertu desquelles les sommes non dépensées à ce titre à compter du 1 janvier 2019 seront reversées.

En effet, l'ensemble des contributions ont vocation à être agrégées par France compétences, puis réparties selon des parts définies par décret. En conséquence, il importe de préciser que toutes les contributions peuvent financer l'intégralité des différents dispositifs. Il convient également d'indiquer que la contribution des entreprises de moins de onze salariés peut financer le compte personnel de formation, comme c'est le cas pour les entreprises de plus de

cause, on diluerait les sommes disponibles pour le financement des autres actions, notamment le développement des compétences dans les très petites entreprises,

Guillotin. Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pénalise les entreprises qui souhaitent embaucher un jeune à l'issue de son contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Ainsi, une entreprise aura davantage intérêt à conclure de nouveaux contrats de professionnalisation ou d'apprentissage qu'à embaucher les jeunes qu'elle vient de recruter en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Nous proposons donc Nous proposons donc que les jeunes embauchés par l'entreprise à l'issue de leur contrat de professionnalisation ou d'apprentissage soient compris dans le quota pendant les trois années suivant l'expiration du contrat en alternance. nous souhaitons permettre aux entreprises de prendre en compte dans leur quota d'alternants les jeunes accueillis en stage obligatoire dans le cadre de leur formation initiale et qui, malheureusement, se heurtent trop souvent à des difficultés pour trouver une entreprise d'accueil.

Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul de cette contribution supplémentaire, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

à la révolution digitale. Il est donc indispensable d'imaginer des modes d'incitation financière permettant le développement des compétences, tout en maintenant une part de mutualisation. Cet amendement vise, d'une part, à renforcer les capacités internes de l'entreprise par un accompagnement de l'opérateur de compétences au titre de la transformation numérique, et, d'autre part, à concrétiser l'incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l'entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l'obligation légale, dont le montant est insuffisant au regard de l'ampleur des besoins. Pour permettre aux TPE et PME de répondre aux besoins en formation

tend à organiser, au sein de l'opérateur de compétences qui sera désigné par la branche, la possibilité de confier la gestion de la contribution à un organisme créé par les organisations représentatives des employeurs et des salariés.

oublié, voire affaibli. Malheureusement, les résultats s'en font déjà sentir. Ainsi, entre 2009 et 2012, le taux de réussite a baissé de sept points, malgré l'instauration d'une épreuve de rattrapage qui permet de repêcher certains élèves. En même temps, entre l'application de la réforme Darcos, donc la réduction d'un an pour la préparation du baccalauréat, la réduction des moyens financiers et le remplacement des remises à niveau dans les matières générales par des heures individuelles sur projet, il n'est pas vraiment étonnant que le nombre de décrochés augmente dans un secteur pourtant de plus en plus considéré comme au seuil d'une révolution. En effet, les métiers agricoles, comme les métiers industriels voilà quelques années, connaissent une période de mutations importantes, avec notamment un nouveau rapport à la production et à la préservation des ressources à mettre en oeuvre.

Malheureusement, et malgré l'opposition des parents d'élève et de l'équipe éducative, il a été décidé que ce dispositif ne serait pas reconduit à la rentrée de septembre 2018, ce qui limite la liberté de choisir leur avenir pour les jeunes du département en situation de handicap. le message envoyé est tout à fait négatif et ne correspond pas à l'objectif que vous nous annoncez depuis le début de l'examen de ce projet de loi, s'agissant notamment des positions que vous avez affirmées, et que je partage,

d'apprentissage et de professionnalisation exercée par les opérateurs de compétences l'est dans le cadre d'une concertation avec les régions. L'objectif est d'éviter la concentration de l'offre de formation en alternance dans les territoires urbains et sur les formations les plus rentables, que de prendre en compte les spécificités territoriales, pour que les CFA des zones rurales ou moins attractives ne soient pas pénalisés et puissent maintenir une offre de formation en direction des jeunes apprentis, notamment ceux qui étudient dans les zones éloignées des métropoles et des grandes villes.

Même avis que la commission. Monsieur Brisson,

cadre des nombreuses auditions que notre groupe a menées pour préparer l'examen du projet de loi, nous avons entendu des représentants des apprentis membres de l'Association nationale des apprentis de France, l'ANAF.

Ils s'inquiètent d'une réduction et de la complexification de l'accès à l'apprentissage pour les jeunes les moins favorisés, aux situations socio-économiques fragiles. La prise en charge de ces aides directes aux apprentis par les régions permettait aussi une adaptation en fonction du contexte local,

Or les apprentis estiment ne pas avoir obtenu de réponse claire du Gouvernement sur ce sujet durant la concertation, non plus que dans le projet de loi. C'est pourquoi nous proposons d'intégrer dans les missions des OPCO le financement des aides directes aux apprentis.

et aucun financement n'est prévu pour les aides directes aux apprentis. En outre, la nature de ces aides et les conditions dans lesquelles elles seraient attribuées ne sont pas précisées. Actuellement, ce sont en effet les régions qui assument.

les niveaux de prise en charge des formations professionnelles. Aujourd'hui, les organismes paritaires collecteurs agréés sont chargés de la gestion et de l'utilisation des fonds de la formation professionnelle et décident des niveaux de prise en charge des formations en fonction des besoins des entreprises, mais aussi

Les branches professionnelles ne sont soumises à aucun cadre national et ne présentent pas forcément de gages d'indépendance vis-à-vis des entreprises. Elles ont de nombreuses missions qui ne leur permettent pas de se spécialiser en matière de formation professionnelle. Selon nous, elles ne sont donc pas habilitées à décider de la prise en charge des formations. Le risque de leur transférer cette compétence est qu'elles jouent sur les niveaux de prise en charge pour orienter les salariés vers certains types de formations.

Dans ce cas, les branches deviendraient un outil à la disposition des employeurs, leur permettant d'adapter les salariés à leurs attentes. Or, pour nous, le choix des salariés en matière de formation professionnelle doit aussi être pris en compte, et ce choix ne peut pas être dicté uniquement par des considérations

: La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis. Cet amendement vise à introduire dans la fixation du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage par les branches des critères complémentaires spécifiques aux régions. Le coût d'un apprenti, à formation équivalente, peut varier très sensiblement selon la région dans laquelle il suit sa formation. L'équilibre financier des CFA ne saurait être garanti par une fixation du coût contrat au niveau national, sans prise en compte des spécificités régionales telles que le prix du foncier, les problématiques de logement ou les écarts salariaux. La fixation par les branches d'un coût au contrat à l'échelle régionale

Votre amendement vise notamment à supprimer les dispositions prévoyant la définition par les branches du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. Outre qu'il ne précise pas comment sera déterminé ce niveau de prise en charge,

469. Madame Delmont-Koropoulis, la commission a précisé les critères qui déterminent la fixation du niveau de prise en charge. Elle a notamment introduit la possibilité de moduler ces niveaux en fonction de critères

fortement à l'échelle nationale, c'est également vrai au sein d'une même région. Je ne suis pas certaine que fixer des critères uniformes pour des CFA se trouvant, par exemple, à Bordeaux

s'élève à 1 000 euros, celui d'une formation débouchant sur un diplôme, à 7 000 euros. Afin que les droits attachés au CPF soient effectifs, il est donc nécessaire d'encourager l'abondement du projet du salarié par l'entreprise, le groupe ou la branche professionnelle. Grace à son service de proximité, l'opérateur de compétences est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise et des branches professionnelles. Il est de ce fait le mieux à même d'inciter l'entreprise, le groupe ou la branche professionnelle à abonder le CPF de ses salariés et d'en faciliter la mise en oeuvre par une gestion unique et simplifiée, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations. Cet amendement vise ainsi un objectif de simplification du circuit financier pour les entreprises, les groupes et branches professionnelles qui souhaitent abonder le CPF de leurs salariés. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter

signe important aux entreprises pour les inciter à financer la formation professionnelle de leurs salariés, au-delà du plan de développement des compétences, dont le financement relève de ces entreprises. Il importe d'encourager les entreprises à dépasser l'intérêt immédiat et à adopter une vision de moyen et long termes. Du fait de sa proximité, l'opérateur de compétences pourra être l'interlocuteur privilégié de l'entreprise et des branches

Le projet de loi prévoit une gestion directe du CPF par la Caisse des dépôts et consignations. Réintroduire un intermédiaire dans certains cas seulement entraînerait une complexification des circuits de paiement qui ne nous paraît pas souhaitable.

lié notamment à des conditions de travail non formatrices, une inadéquation à la formation suivie ou des exigences de productivité ne correspondant pas à ce que doit être l'engagement d'un apprenti, est repéré

Au contraire, dans une logique de responsabilisation et de liberté d'initiative, il me semble souhaitable de laisser les partenaires sociaux décider au sein de chaque organisme des actions que ceux-ci souhaitent mettre en oeuvre au service des employeurs

M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à préciser que les conventions d'objectifs et de moyens entre l'État et les opérateurs de compétences ont vocation à être évaluées dans des conditions déterminées par décret. En effet, cette évaluation incombe

entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés et entreprises de 300 salariés et plus. Le projet de loi supprime ces sous-sections au profit d'une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés seraient donc regroupées au sein d'une même et unique section comptable, ce qui pourrait s'avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE. En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais aussi de la rémunération du salarié en formation, ainsi que des frais annexes. Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser plus spécifiquement les entreprises de 11 à 49 salariés, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation, et ainsi d'assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés. C'est pourquoi il paraît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés,

en limitant les ressources consacrées aux entreprises de moins de 11 salariés. Il faudrait par ailleurs prévoir des règles d'affectation des fonds entre ces deux sous-sections.

poursuivez. Aujourd'hui, même si les entreprises de moins de 11 salariés et de 11 à moins de 50 salariés bénéficient d'une sous-section particulière, il apparaît que la mutualisation pour les entreprises de plus petite taille est non seulement inefficace, mais se fait au détriment de ces dernières. En effet, en 2016, les entreprises de moins de 11 salariés n'ont bénéficié au titre de la mutualisation que de 5,8 millions d'euros venant des entreprises de plus de 50 salariés, contre 15,3 millions pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés. Cette relative faiblesse s'explique par le fait que seules les entreprises de moins de 300 salariés contribuaient au plan de formation. Pour le dire de

C'est pourquoi le nouveau système, qui oblige non plus simplement les petites et moyennes entreprises, mais toutes les entreprises à participer à l'effort de mutualisation en faveur des plus petites entreprises me semble pouvoir davantage répondre à leurs besoins. Par ailleurs, le développement de la formation dans les TPE-PME est l'une des missions des OPCO et fera l'objet d'un suivi attentif

Il est proposé de rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale en matière de définition du niveau de prise en charge des coûts des CFA ainsi que des frais annexes à la formation des apprentis relevant de l'intervention de l'opérateur de compétences. En effet, il importe de poursuivre les travaux avec les réseaux de CFA afin de définir par voie réglementaire de manière plus fine le périmètre du financement au contrat. l'accompagnement du salarié en amont de la signature de son contrat pourrait dépendre demain davantage d'un financement relevant de la préparation à l'apprentissage couvert par le plan d'investissement dans les compétences, soit par un autre circuit financier que les fonds de l'alternance dédiés au financement des salariés en contrat. Par ailleurs, il appartiendra plutôt aux régions de déterminer les majorations du financement au contrat qu'elles estiment pertinentes en fonction de besoins d'aménagement du territoire c'est dans ce cadre que des surcoûts liés à l'implantation dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone rurale pourront être compensés, en fonction de spécificités territoriales naturellement différentes d'une région à une autre. Enfin, les frais annexes à la formation des apprentis visent les dépenses de restauration et d'hébergement nécessaires à l'attractivité des CFA et au développement de ce type de formation. Le coût du foncier a plutôt vocation à être intégré comme un déterminant du niveau de prise en charge au contrat. L'amortissement des investissements réalisés, quand il s'agit d'équipements pédagogiques notamment, gagne à être pris en compte dans le financement au contrat. C'est la philosophie globale du financement de l'apprentissage tel que refondé par ce projet de loi que nous souhaitons donc rétablir.

Il est proposé que la base de calcul du coût par apprenti soit la plus complète possible, s'alignant ainsi sur les coûts réellement supportés par les CFA. Le présent amendement vise, d'une part, à préciser les éléments servant de base au calcul du coût au contrat et, d'autre part, à intégrer la taille de l'entreprise signataire du contrat d'apprentissage dans les critères de modulation du niveau de prise en charge défini par les branches professionnelles.

Il s'agissait en l'occurrence de s'assurer que les différents déterminants économiques et géographiques, notamment les coûts exposés par les centres de formation des apprentis, seraient bien pris en compte. Les auteurs de l'amendement renvoient à des travaux qui doivent être menés avec les CFA. Il me semble qu'il aurait été pertinent de mener de tels travaux avant de légiférer. La commission estimant que le texte résultant de ses travaux offre les garanties nécessaires, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

devront ainsi être pris en compte les coûts spécifiques à chaque formation, l'accompagnement des salariés en amont du contrat et des salariés résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, les frais liés au coût du foncier, à l'amortissement des investissements et à l'aide au transport. Tous les critères ne pouvant être inscrits dans la loi, il s'agit de prévoir un socle minimal.

Les petites entreprises sont en effet les principales formatrices des apprentis et il ne faut pas qu'elles soient freinées dans leur embauche. Les autres critères proposés sont satisfaits. La modulation en fonction des financements publics peut être utile pour les formations en apprentissage hébergées par des établissements d'enseignement.

l'accompagnement des salariés en amont du contrat et des salariés résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, les frais liés au coût du foncier, à l'amortissement des investissements et à l'aide au transport.

un impact sur l'intérêt du jeune et sur le fonctionnement du centre de formation ? Il me semble que non.

Avec la réforme, les régions vont bénéficier d'une dotation visant à apporter un concours financier aux CFA, dont le financement au contrat ne permettra pas d'assurer l'ouverture, voire le maintien de certaines sections d'apprentissage en sous-effectif. En pratique, les régions vont recevoir une enveloppe de 250 millions d'euros pour aider les CFA en difficulté, et une autre au titre de l'investissement à hauteur de 180 millions d'euros.

pour prendre en compte le fait que certaines formations en apprentissage sont hébergées dans des établissements de l'éducation nationale. La commission a donc émis un avis défavorable.

vise à pérenniser le financement de la formation des bénéficiaires de la préparation opérationnelle à l'emploi, qui permet à un jeune ou à un demandeur d'emploi d'acquérir les prérequis qui lui font défaut pour répondre à une offre d'emploi. Ce dispositif bénéficie d'un financement partiel de Pôle emploi qui intervient sur la rémunération du stagiaire et sur une partie du coût de la formation.

au titre des CFA ou de l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Si tel devait néanmoins être le cas, l'enveloppe financière dont ils disposent n'étant pas extensible, la prise en charge du salaire des apprentis se ferait au détriment des autres missions des OPCO. L'avis est donc défavorable.

Cet amendement vise à rendre éligibles les actions de formation des salariés de l'insertion par l'activité économique, l'IAE, aux financements de l'alternance, permettant aux structures d'accéder à des financements à hauteur de leurs besoins et capacités et traduisant que l'IAE constitue dans son fonctionnement actuel une forme d'alternance adaptée pour les personnes très éloignées de l'emploi.

à Mme la ministre. Cet amendement vise à permettre aux opérateurs de compétences d'accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle lorsqu'ils financent des formations pour les demandeurs d'emploi. Les opérateurs de compétences pourront ainsi accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle

Savary. Cet amendement vise à obliger les seules branches professionnelles souhaitant changer d'opérateur de compétences au 1 janvier 2019 à négocier un accord de désignation d'opérateur de compétences avant le 31 octobre 2018.

? Ces amendements prévoient que, pour les branches qui le souhaitent, l'OPCA aujourd'hui habilité devienne un OPCO sans qu'un nouvel accord soit nécessaire. Il me semble juridiquement fragile de prévoir un transfert de l'agrément d'un OPCA qui cesse d'exister d'exister à un OPCO, qui doit juridiquement être une nouvelle structure, d'autant que l'alinéa 102 précise que les agréments perdront leur validité au 1 avril 2019

en ce qu'il s'exerce sur le domaine public, est, plus que d'autres, encadré et réglementé dans son accès et son exercice d'activité. Ces spécificités ont conduit le secteur à mettre en place un organisme compétent et opérant dans le développement de la formation professionnelle, lequel exerce déjà ses missions de manière complémentaire avec l'actuel OPCA. Cet amendement prévoit que le futur opérateur de compétences exerçant dans le secteur des transports peut conclure une convention avec l'organisme visé à l'article 1635 M du code général des impôts, lequel possède les compétences requises pour permettre le développement de la formation professionnelle dans le domaine des transports. Cette convention définit les conditions de leur coopération et de répartition des missions. Toutefois, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement afin de savoir si une telle convention n'est pas possible sans une disposition législative spécifique.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L'article 20 habilite le Gouvernement à fixer par ordonnances dans un délai de dix-huit mois les mesures afin d'attribuer aux URSSAF le recouvrement, l'affectation et le contrôle des contributions des employeurs destinées au financement de la formation professionnelle. Cet article prévoit également l'habilitation du Gouvernement d'harmoniser l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ainsi que d'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet. Notre groupe est opposé à la pratique des ordonnances dans la mesure où le dessaisissement du du Parlement l'affaiblit considérablement au profit du Gouvernement, déséquilibrant davantage encore les institutions de notre République. En prévision de nos futurs échanges sur la réforme de la Constitution, nous ne pouvons que déplorer la démultiplication du recours aux ordonnances. Pour cette raison, nous demandons la suppression de l'article 20. Quel ? Nous avons adopté l'article 17, qui prévoit une réforme de la contribution au financement de la formation professionnelle ainsi que de la taxe d'apprentissage. Il est prévu que ces impositions seront à l'avenir collectées par le réseau de l'URSSAF. L'ordonnance prévue par le présent article est

en supprimant de son champ le transfert du recouvrement, de l'affectation et du contrôle de la contribution au développement des formations professionnalisantes, qui est versée directement par les entreprises aux établissements de formation initiale et technologique et aux organismes éligibles fixés à l'article 17 du projet de loi. inclut dans le champ de l'ordonnance la possibilité de procéder à des ajustements législatifs liés à la collecte, l'affectation aux branches concernées et le contrôle du bon recouvrement des contributions conventionnelles, décidées librement par les branches, afin de permettre leur usage sécurisé de l'URSSAF, dans des modalités à déterminer. Ces contributions conventionnelles relèvent du champ de la formation professionnelle ou du développement du dialogue social. ? Cet amendement vise à étendre le champ d'une habilitation demandée par le Gouvernement. Or, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les parlementaires ne peuvent être à l'origine ni d'une habilitation à légiférer par ordonnances ni de l'extension du champ d'une habilitation demandée par le Gouvernement. Tout à fait ! Je vous propose donc, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond, de déclarer cet amendement contraire à la Constitution.

qui, comme le principe même de l'habilitation l'implique, doit émaner du Gouvernement. Sous votre contrôle, madame la présidente, et sous celui des sachants du service de la séance, rien ne s'oppose à ce que Mme la ministre reprenne cet amendement.

conduirait les entreprises à percevoir ces contributions volontaires comme des prélèvements obligatoires et non comme des démarches volontaires d'adhésion.

Mme la rapporteur. Je vous prie de m'excuser, madame la ministre, mais les contributions supplémentaires sont à la fois les contributions volontaires et les

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement concerne une nécessaire adaptation territoriale pour les collectivités concernées. En effet, le transfert de la gestion des CFA aux branches professionnelles est dangereux pour l'avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d'être où, faute d'être suffisamment structurées, elles sont incapables d'assumer seules cette compétence. La taille réduite des territoires et le volume limité des publics pouvant y être accueillis contribueront à ce que les centres de formation des apprentis ne soient pas à même de remplir des objectifs fixés au niveau national. La valorisation du compte personnel du salarié en euros n'est pas adaptée aux coûts unitaires moyens complets des formations financées. Le différentiel de coût horaire est de l'ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l'Hexagone. Enfin, dans certains territoires, le financement de la formation fait peser des risques sur le statut juridique et la pérennité de certains établissements

qui a proposé lors de l'audition de la ministre en commission, puis dans le cadre de la délégation aux outre-mer d'identifier les adaptations nécessaires, nous pousse aujourd'hui à proposer des amendements collant à la réalité et aux besoins de nos territoires ultramarins. Quel ? Compte tenu de la situation outre-mer, il s'agit d'un ajout utile. Les collectivités concernées doivent pouvoir être consultées sur le décret prévoyant les modalités d'application dans les départements des règles relatives à la formation professionnelle. En conséquence, l'avis est favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Je comprends et je partage, comme vous le savez, votre point de vue sur la nécessité d'associer étroitement les différents acteurs ultramarins au processus d'élaboration des normes

déjà une consultation obligatoire des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative

Cet amendement rédactionnel tend à procéder à un changement de références en raison de la modification de l'article 17 relatif au financement de la formation professionnelle.

par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues par l'article L. 1442-5 du code du travail. En effet, l'abrogation du système de dépense libératoire prévu à l'ancien article L. 6331-1 du code du travail rend impossible la compensation des salaires maintenus pour leurs salariés qui s'absentent de leur entreprise dans le cadre de leur formation initiale obligatoire. Cet amendement vise à supprimer la référence à cet article aujourd'hui abrogé et à préciser que les jours de formation initiale font l'objet d'une indemnisation au titre des activités prud'homales. À cet

elle couvre la formation initiale et continue. Aussi, nous avons du mal à mesurer l'intérêt de la précision apportée au travers de cet amendement, qui vise l'obligation par l'employeur d'accorder au salarié le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales. En conséquence, nous émettons un avis de sagesse, et j'aimerais connaître

Il est préférable de procéder à chaque remplacement nécessaire en visant tous les articles concernés. Le texte prévoit que le Gouvernement sera habilité par ordonnance à prendre les mesures de coordination nécessaires. Absolument ! En conséquence,

Dans le cadre de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a confirmé sa volonté d'aider les départements et les collectivités d'outre-mer dans la recherche de solutions pérennes au développement de l'offre de formation. Cet amendement s'inscrit dans la même démarche, en demandant la remise d'un rapport d'information au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la loi. Celui-ci aura comme objet de chiffrer les surcoûts de formation pour les personnes issues des territoires ultramarins, afin de faire un état des lieux de l'offre de formation, tout en identifiant les problèmes liés à la mobilité des personnes dans les territoires qui entraînent de fait des coûts supplémentaires. D'une part, ce rapport permettra une meilleure concertation entre les parlementaires et le Gouvernement et, d'autre part, il servira de base solide à la rédaction des ordonnances spécifiques à l'outre-mer que le Gouvernement sera habilité à prendre au travers de l'article 66 du projet de loi.

France compétences a pour mission d'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle. Les territoires ultramarins sont bien sûr couverts par cette mission et ils bénéficieront d'une attention particulière au regard de leurs spécificités. Dans ces conditions, il ne me semble pas nécessaire de prévoir un rapport d'information spécifique sur ce sujet. Aussi, je propose le retrait

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur dès la promulgation de la loi des dispositions de l'article 8 afin de faciliter l'accès à l'apprentissage des mineurs qui seront amenés à effectuer, dans le cadre de leur formation, des périodes d'emploi ou de stage dans des débits de boissons sans être affectés au service du bar. C'est le cas, par exemple, des jeunes qui seront strictement affectés à la réception ou au service des chambres dans le cadre de leur formation pratique.

Tout d'abord, je veux saluer l'initiative des députés concernant l'ajout de cet article, qui prévoit l'allongement de la durée maximale du premier contrat de professionnalisation de trois à cinq ans entre les jeunes sportifs et le club formateur ; c'est une très bonne chose. Vous me voyez inspirée, car je reviens juste du département de Meurthe-et-Moselle où, avec la ministre

Une partie d'entre eux seront amenés à entamer et à réussir une brillante carrière sportive professionnelle, à l'instar des joueurs de l'Équipe de France, qu'il convient ici collectivement, me semble-t-il, de féliciter et, surtout, d'encourager pour la finale de dimanche prochain. Il est en effet opportun de donner aux clubs tous les moyens de bâtir des effectifs solides, reposant sur un système de formation équilibré et s'inscrivant dans la durée et dans l'intérêt non seulement du sport et des fédérations, mais, surtout, également des jeunes athlètes. Avec cette disposition, le sportif se verra proposer un contrat d'une durée de cinq ans, contre trois ans auparavant, un gage de confiance et de sérénité, conditions nécessaires à la progression et à la performance. Cette disposition louable vise en même temps à protéger les jeunes joueurs, à assurer nos fédérations d'un vivier de jeunes talents,

La relation entre le club employeur et le joueur salarié justifie de fait le renvoi au dialogue social, qui apparaît nécessaire pour protéger les jeunes joueurs et leur faire bénéficier d'un encadrement adapté. Les clubs pourront ainsi s'investir davantage.

L'article 25 A a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement. Je note toutefois que son lien avec le projet de loi n'est qu'indirect, puisque nous abordons la question des jeunes sportifs professionnels,

Cet article porte de trois à cinq ans la durée maximale du premier contrat qu'un sportif peut être obligé de signer avec le club qui l'a formé, alignant ainsi la durée maximale de ce premier contrat sur la durée maximale des contrats de sportif professionnel. qui a créé cet article a suscité de nombreuses réactions dans le monde du sport, un certain nombre d'acteurs considérant que le Gouvernement et sa majorité profitaient de l'examen de ce texte sur la formation professionnelle pour court-circuiter des négociations en cours. Je ne peux m'empêcher de faire remarquer que, lorsque l'on ajoute en cours de discussion des dispositions qui n'ont pas été préparées et qui n'ont pas fait l'objet de négociations ou des concertations nécessaires, on s'expose inévitablement à ce type de critiques. S'agissant de l'amendement n° 152 rectifié, il est apparu à la commission que la durée maximale prévue par le code du sport ne faisait pas obstacle à ce qu'une convention collective particulière prévoit une durée inférieure en cas d'accord en ce sens entre les partenaires sociaux. Ainsi, si les partenaires sociaux du football, puisqu'il s'agit principalement de ce sport, mais aussi de tout autre sport professionnel, décidaient de maintenir, dans leur charte, une durée maximale de trois ans, ils en auraient

? Le Gouvernement est favorable à l'amendement, parce que l'appréciation de la durée idoine du contrat de futur joueur professionnel, qui termine son cycle de formation, nécessite une certaine souplesse, ainsi que la prise en compte des spécificités de certains sports et de certaines organisations dans certaines fédérations. En outre, je pense que le fait de renvoyer au dialogue social sectoriel permettra de mieux prendre en compte les spécificités de chacune des disciplines structurées professionnellement et les situations particulières des clubs employeurs,

depuis 2014. Cette situation est pénalisante et aurait dû faire l'objet d'un rapport du Gouvernement au titre de l'article 16 de la loi du 1mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

Depuis 2014, les centres de formation des clubs professionnels ne sont plus éligibles à la perception de la taxe d'apprentissage. Or ces centres accueillent des jeunes à partir de quinze ans qui, en parallèle de leur formation professionnelle de footballeur, suivent des parcours scolaires professionnalisants. Cet amendement vise à reconnaître la qualité de CFA à ces centres. Cela permettra également aux élèves de bénéficier, de fait, du statut d'apprenti. Je rappelle que la France compte aujourd'hui 4 800 sportifs sous convention de formation.

Les règles qui les concernent sont distinctes et les jeunes sportifs de haut niveau ne sont pas des apprentis. Il ne serait donc pas pertinent que les financements dédiés à l'apprentissage soient versés aux centres de formation sportifs. De plus, comme les fonds destinés aux CFA relèvent d'une enveloppe fermée, cette extension entraînerait une dilution des financements dont bénéficient les CFA aujourd'hui.

les jeunes qui sont dans les centres de formation des clubs sportifs ne se préparent pas tous à des métiers ou à des diplômes relevant du ministère des sports, ce qui pénalise

des centres de formation des sportifs. D'ailleurs, il faut rappeler que, pour ceux qui figurent sur la liste des sportifs de haut niveau, qui dépend du ministère des sports, ce rapport était d'ores et déjà prévu dans la loi dite « Braillard » du 1mars 2017 du 1mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. Ce rapport devait être remis

prévoit que les contrats de travail, de même que les contrats de prestation de services, les contrats de cession de droit à l'image ou les contrats de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge, peuvent donner lieu à la signature d'une convention-cadre avec l'État. Il conviendrait ici d'inclure les contrats d'apprentissage et les contrats professionnels pour sécuriser la compensation offerte aux entreprises mettant en place ce type de conventions, adaptées aux emplois du temps et contraintes des sportifs de haut niveau qui

Je vais encore me répéter, parce qu'il existe, selon moi, une évidence légale sur le sujet : les contrats d'apprentissage et les contrats professionnels sont des contrats de travail.

Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à zéro heure trente environ, afin d'aller plus avant dans l'examen de ce texte.

amendement. Celui-ci vise en effet à récrire l'article 33 du projet de loi, afin de confier aux partenaires sociaux le soin de négocier de nouveaux accords d'assurance chômage sans attendre l'échéance de l'actuelle convention, qui est fixée au mois de septembre 2020. Cette négociation se fera sur la base d'un document de cadrage, soumis à la concertation préalable des partenaires sociaux. Elle visera notamment à faire évoluer les règles actuelles pour mieux lutter contre la précarité de l'emploi, inciter les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi, et revoir l'articulation entre assurance et solidarité. Alors, pourquoi cet amendement ? ? Premièrement, l'amendement vise à tenir compte des différentes remarques formulées aussi bien par les députés que par les sénateurs, mais aussi par les partenaires sociaux, sur le projet initial du Gouvernement qui tend à déterminer par décret certaines des règles de l'assurance chômage au regard des adaptations jugées nécessaires,

par le Président de la République devant le Congrès, cet amendement s'inscrit dans la volonté présidentielle de refonder la politique contractuelle, en s'appuyant sur les partenaires sociaux, tout en menant à bien les transformations nécessaires pour conjuguer progrès économique et progrès social. le Gouvernement entend assurer une mise en oeuvre rapide et efficace de la réforme de l'assurance chômage, notamment en ce qui concerne la lutte contre la précarité et la permittence, tout en ouvrant la possibilité aux partenaires sociaux de mieux prendre en compte le chômage de longue durée dans l'indemnisation des demandeurs d'emploi.

social élargi avec l'État. Dans le cadre de cet agenda social plus large, dont le contenu sera débattu dans quelques jours entre le Président de la République et les partenaires sociaux, il importe que l'ensemble des champs importants soient ouverts et puissent être ouverts à la négociation. C'est le cas notamment de l'assurance chômage. Voilà les trois raisons pour lesquelles je vous invite à adopter cet amendement.

S'agissant de la méthode, il n'est pas acceptable qu'un amendement aussi important soit déposé aussi tardivement. Notre commission ne dispose sur cette mesure ni d'étude d'impact, ni de l'avis du Conseil d'État, ni du temps suffisant pour organiser des auditions complémentaires. Alors que le Gouvernement envisage une réforme institutionnelle qui remet en cause les prérogatives du Parlement, nous avons entendu lundi dernier le Président de la République annoncer le dépôt d'un amendement pour ouvrir de manière anticipée les négociations sur la convention d'assurance chômage. Ce n'est pas la conception que nous nous faisons de relations sereines entre le Parlement et le Gouvernement. La majorité des responsables des groupes politiques au Sénat a manifesté mardi sa réprobation à l'égard de la méthode employée par le Gouvernement. je vous rappelle que la méthode retenue pour élaborer ce projet de loi est contestable, car plusieurs sujets ont été introduits tardivement, comme l'emploi des travailleurs handicapés, les plateformes numériques, tandis que les dispositions relatives aux travailleurs détachés ne semblent toujours pas stabilisées. Sur le fond, l'amendement pose quatre difficultés.

le Conseil constitutionnel a jugé qu'une loi ne saurait porter une atteinte excessive à des accords collectifs antérieurs, légalement conclus, sauf motif d'intérêt général suffisant. En effet, « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles IV et XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. L'amendement ne démontre pas pour l'instant un intérêt général suffisant. Ensuite, l'amendement ne prévoit pas explicitement que la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et ses textes associés deviendront caducs. L'amendement porte sur le futur, mais ne règle pas la situation actuelle.

Enfin, l'amendement prévoit que le document de cadrage proposera aux partenaires sociaux de revoir l'articulation entre les allocations chômage assurantielles et celles de solidarité. on ignore à partir de quand la nouvelle allocation de chômage longue durée pourrait être accordée : deux ans ou plus pour les seniors ? Ce faisant, l'amendement brouille un peu plus la frontière entre ces deux allocations. On ne peut pas à la cantonade modifier ainsi des principes historiques de la protection sociale sans une vision globale et un temps de réflexion nécessaire. Le Conseil d'État, dans son avis sur le texte, a souligné l'importance d'une vision globale pour réformer la protection sociale : « Le Conseil d'État invite le Gouvernement à approfondir sa réflexion sur la cohérence des modalités de financement des régimes avec les prestations qu'ils servent, dans la perspective d'une réforme du système de protection sociale ».

de la méthode employée par le Gouvernement- elle a déjà été dénoncée lors de nombreux rappels au règlement sur l'ensemble de nos travées -, le projet de loi instaure la mainmise de l'État sur l'assurance chômage sous plusieurs aspects. D'abord, le texte donne le contrôle des finances à l'État, en remplaçant le financement par les cotisations sociales par un financement par l'impôt. Ce n'est pas anodin ; c'est même lourd de conséquences. Ensuite, il dessaisit les partenaires sociaux de leur capacité de négocier.

Lorsque le Gouvernement annonce vouloir renégocier immédiatement la convention d'assurance chômage, normalement en vigueur jusqu'en 2019, afin d'ouvrir l'allocation chômage au-delà de vingt-quatre mois, c'est de la poudre aux yeux L'objectif d'une telle mesure est uniquement de pouvoir négocier la convention selon les nouvelles règles issues du projet de loi, ce qui permettrait au Gouvernement de prendre définitivement le contrôle sur l'assurance chômage.

c'était un dégrèvement- c'est ce qui nous avait été présenté en commission. Mais cela justifie-t-il de changer tout l'équilibre de la protection sociale ?

Il est tout à fait possible- cela nous arrive à tout moment dans la vie parlementaire -de regretter les conditions d'arrivée d'une proposition dans un débat.

respect un certain nombre de critiques sur les prises de position unilatérales, directives, du Gouvernement, qui ne tiendrait pas suffisamment compte des appréciations et du poids des partenaires sociaux. En on corrige un dispositif législatif en cours en tenant compte des événements récents de la vie sociale que Mme la ministre a mentionnés pour rouvrir- à mon sens, beaucoup des partenaires sociaux sont intéressés par cela et ne demandent pas de délai supplémentaire ; ils préfèrent que l'on travaille tout de suite -un champ à la négociation sociale sur des enjeux majeurs, dont, si j'ai bien compris, personne ne conteste le caractère décisif. Il s'agit de la multiplication des contrats courts, y compris dans une période de reprise de l'emploi, et de la persistance d'un chômage structurel, qu'il est difficile de traiter dans la durée.

tout à l'heure. Plusieurs des objections qui ont été élevées par la rapporteur Puissat sont surmontables. Madame, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté contractuelle remplit quelques volumes. Elle consiste toujours à à reconnaître l'importance d'un motif d'intérêt général qui vient limiter la liberté contractuelle, spécialement entre les partenaires sociaux. Si vous voulez soutenir que la lutte contre les contrats courts et l'action contre le chômage structurel ne sont pas des motifs d'intérêt général suffisants, c'est une ascension de la face nord ! J'en viens au sujet de fond.

des questions que je me pose. Pourquoi prendre le risque d'inconstitutionnalité ? Pourquoi prendre le risque de bousculer les procédures admises habituelles Pourquoi prendre le risque d'une manifestation de mépris à l'égard du Parlement ? Pourquoi prendre le risque de remettre en cause tout le travail de réflexion, d'élaboration d'amendements et de débat Pourquoi laisser prendre autant le risque d'apparaître comme totalement amateurs et montrer l'impréparation de votre texte ? texte ? Contrairement à ce que vous avez dit, madame la ministre, ce n'est pas une mince affaire ! Il ne s'agit pas simplement de regarder si l'on peut moduler le cumul entre emploi partiel et allocations. Non ! Le Président de la République a déclaré qu'on allait confier aux partenaires sociaux le soin de réviser les règles de l'assurance chômage ; il a même évoqué la « transformation de l'assurance chômage

Quelques rappels cependant sur la gouvernance de l'assurance chômage. Qu'en est-il actuellement ? La loi délègue aux partenaires sociaux la définition des règles d'indemnisation par la voie conventionnelle. Nous ne sommes pas pour autant dans une pure gestion paritaire, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, le Gouvernement n'est jamais bien loin pour faire valoir son point de vue, articuler ses propres interventions avec celles de l'UNEDIC et servir d'instance d'appel sur les sujets difficiles il faut bien que se tienne le festival d'Avignon ! Rappelons que le Gouvernement agrée la convention d'assurance chômage. Il est donc bien, à la différence du Parlement, l'un des acteurs principaux du scénario actuel. Deuxièmement, le recours à l'endettement ne sert pas seulement d'ajustement aux aléas de la conjoncture. Il offre également une porte de sortie commode aux négociateurs pour le bouclage des conventions. La proposition du Gouvernement fait évoluer ce schéma de gouvernance : un document de cadrage fixera désormais le cap de la négociation. En supprimant les contributions salariales et en créant une aide forfaitaire pour les travailleurs indépendants, le Gouvernement fait évoluer la nature de l'indemnisation du chômage vers des prestations de solidarité. En mettant fin par anticipation à l'actuelle convention, valide jusqu'en 2020, dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas très claires, le Gouvernement demande paradoxalement aux partenaires sociaux d'acter cette évolution dans une nouvelle convention négociée dans le nouveau cadre et reverrait à cette occasion les règles des allocations de solidarité. Nous assistons à la dépossession des partenaires sociaux des prérogatives qui leur ont été déléguées par la loi, à travers la remise en cause des accords conclus. Comme vient de le rappeler notre rapporteur Frédérique Puissat, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 août 2008 sur la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a fixé la doctrine en pareil cas : une convention ne peut être remise en cause par le législateur que pour un motif d'intérêt général suffisant. Quel est le motif d'intérêt général suffisant que le Gouvernement entend invoquer pour remettre en cause une convention agréée voilà un peu plus d'un an ? C'est la question que nous posons au Gouvernement. Nous demanderons évidemment au Conseil constitutionnel d'examiner sa réponse.

en présentant une cohérence : construire « l'État-providence du XXI siècle ». Ce qui semble être une formule nouvelle est en réalité une formule déjà éculée depuis la fin du siècle dernier par certains qui ont essayé de revenir sur notre modèle, y compris dans d'autres pays européens.

». La responsabilité passe par l'acceptation accrue des postes, quels qu'ils soient, par les chômeurs. En cela, le système qui est proposé est fort commode, avec son financement par l'impôt. Il évacue les partenaires sociaux et permet à l'État d'imposer ses conditions aux chômeurs. C'est effectivement cohérent avec la volonté d'orienter de plus en plus de personnels de Pôle emploi vers le contrôle des chômeurs, alors que les besoins en termes d'accompagnement, notamment des chômeurs de longue durée,

Je reviendrai maintenant sur le motif d'intérêt général, puisque vous m'avez interpellée sur ce sujet. Pour nous, il y a un motif d'intérêt général important qui justifie de demander au législateur d'anticiper

à trois enjeux extrêmement importants. Le premier enjeu, qui est croissant, c'est la lutte contre la précarité excessive. Comme vous le savez, 80 % à 85 % des embauches se font aujourd'hui en CDD,

qui ne se justifie pas et qui a besoin d'être régulée. C'est un motif d'intérêt général extrêmement important. Comment peut-on

juste une chose : autoriser les partenaires sociaux à renégocier des éléments de la convention d'assurance chômage. C'est aussi par respect du dialogue social que nous considérons que le fait d'élargir le champ leur permettra de choisir les bons leviers et d'en négocier entre eux.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande Le scrutin est ouvert.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

Cet amendement vise à supprimer la possibilité que s'octroie le Gouvernement de modifier les règles d'indemnisation des chômeurs

pour deux raisons. La première raison, c'est que l'alinéa 1 autorise le Gouvernement à fixer par décret les règles de l'allocation des démissionnaires et des travailleurs indépendants afin de garantir l'effectivité de ces deux nouvelles allocations, disposition que nous n'avons pas encore votée mais que nous avons présentée en commission. La seconde raison, c'est que je souhaite donner un délai supplémentaire aux branches pour négocier sur la précarité. C'est ce que nous verrons demain matin.

supprimer la disposition permettant au Gouvernement de déterminer par décret les conditions dans lesquelles l'allocation chômage des travailleurs indépendants peut se cumuler avec les revenus d'activité et les revenus sociaux. La question du cumul des revenus est une question sensible, car elle concerne les personnes les plus fragiles économiquement et socialement. socialement. C'est ce cumul de revenus qui permet aux foyers les plus précaires de tenir financièrement. Si cette question est centrale pour les travailleurs salariés, elle l'est encore plus pour les travailleurs indépendants. En effet, pour l'instant, cette catégorie de travailleurs ne bénéficie pas d'une assurance chômage. Ce projet de loi prévoit de leur ouvrir ce droit, mais de façon restreinte par rapport à l'allocation chômage des salariés. Selon les annonces du Gouvernement, l'allocation chômage serait de 800 euros par mois pendant six mois maximum. Cette allocation est faible puisqu'elle est inférieure au seuil de pauvreté estimé par l'INSEE à 1 000 euros par mois. Il est donc crucial pour ces travailleurs indépendants de pouvoir cumuler l'allocation chômage avec des revenus de leur travail plus ponctuels. Cette question du cumul de revenu est essentielle et doit donc être débattue au sein du Parlement et non dans le cadre de l'article 38. Quel est l'avis de la commission ? La commission a

Ensuite, le décret visé au premier alinéa de l'article 33 a une portée très limitée, essentiellement technique, pour permettre la mise en place de l'allocation des travailleurs salariés. Comme vous le savez, j'ai un regard plutôt critique sur cette allocation, mais à partir du moment où elle existera, il faudra des textes d'application pour la faire vivre.